d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Mme Agnès Canayer,

qui a cours sur l'une des mers les plus fréquentées au monde, est au coeur de la relation franco-britannique. Indépendamment du transport de marchandises, le trafic des voyageurs représente une activité essentielle pour nos territoires littoraux. Or, depuis plusieurs mois, le trafic transmanche de voyageurs traverse une crise inédite. En mars dernier, la compagnie P&O Ferries a licencié, à distance et par surprise, 800 de ses marins, qui ont été remplacés par des travailleurs non européens à très bas salaires et soumis à de fortes amplitudes horaires.

qui d'autres qu'eux pour assurer la surveillance de nos massifs et des espèces qu'ils abritent ? Cette question est d'autant plus impérieuse que certaines de ces maisons forestières, à l'instar de celle de Guermange, en Moselle, se situent dans des sites protégés Natura 2000 Natura 2000 ou classés « réserves de biosphère » par l'Unesco. Les économies financières résultant de la fermeture des maisons forestières dans ces sites ont en réalité un coût exorbitant : la disparition des espèces, voire des forêts elles-mêmes Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour freiner ces fermetures et ce désengagement de l'État dans la protection de nos forêts et de leur écosystème ?

vous remercier de votre engagement en faveur des forêts et m'associer au soutien que vous avez exprimé en faveur de nos forces de sécurité civile, en particulier de nos sapeurs-pompiers, qui ont fait preuve d'un courage et d'une abnégation

prochain décret autorisant la cession d'immeubles bâtis domaniaux. Je précise que, grâce à la gestion sylvicole exemplaire de ce massif forestier, une espèce protégée est réapparue : le rapace appelé pygargue à queue blanche. Dans le cadre de la stratégie immobilière fixée par l'État, l'ONF a défini un parc de logements à conserver pour plusieurs raisons,

à cette situation des réponses adéquates. Bien entendu, la France doit accentuer ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais le changement climatique est d'ores et déjà une réalité et il n'y aura pas de retour en arrière. La ressource en eau représente donc un enjeu crucial. Quel avenir pour l'oignon doux des Cévennes, production emblématique du territoire, sans un accès à l'eau ? Il nous faut renforcer la résilience de l'agriculture française, tout en évitant les conflits d'usage. Cela passera par l'adaptation des pratiques agricoles, mais également par des investissements permettant de sécuriser l'accès à la ressource. Les retenues collinaires, qui permettent de stocker l'eau lors des saisons plus humides pour la prélever lors des saisons sèches, peuvent s'avérer pertinentes et efficaces dans certains territoires.

de telles dispositions semblent relever du bon sens. Monsieur le secrétaire d'État, quelles dispositions comptez-vous prendre pour favoriser et accélérer la réalisation de ces ouvrages lorsqu'ils s'avèrent pertinents et ne menacent pas les écosystèmes aquatiques ? La

Fesneau. Je le sais, l'accès à la ressource en eau est un sujet important pour vous et la gestion de cette ressource représente un enjeu crucial pour un département magnifique comme celui du Gard. Vous le savez mieux que moi, monsieur le sénateur, il n'y a pas d'agriculture ni d'alimentation sans eau. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un enjeu de souveraineté alimentaire ; je viens d'ailleurs moi-même d'un territoire, les Côtes-d'Armor, qui est important pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Votre constat est donc pleinement partagé par le Gouvernement, monsieur le sénateur. C'est pour y répondre que nous avons lancé, en 2021, le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. C'est une feuille de route qui doit nous permettre de répondre aux enjeux liés à l'eau, dans un contexte de dérèglement et de changement climatiques auquel sont confrontés l'agriculture et nos agriculteurs. Dans le cadre de cette dynamique, nous travaillons dans plusieurs directions, pour améliorer notre capacité à stocker l'eau quand elle est en excès afin de pouvoir l'utiliser lorsque les agriculteurs en ont le plus besoin.

Mon collègue Marc Fesneau procède chaque semaine, en lien avec tous les préfets concernés, à une revue des projets, région par région. Cela permet, territoire par territoire, de simplifier, d'accélérer, de faciliter les projets déjà bien ficelés ou prêts. Il faut le faire de manière concertée, en lien avec vous, les élus, et dans le respect de nos engagements environnementaux. Cette revue des projets permet également d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées localement et de faire en sorte que, là où il y a des blocages, nous puissions y remédier.

terminer leur plan d'adaptation, de même que les chambres d'agriculture. Cela permettra d'analyser la dynamique des acteurs des filières, pour déterminer les besoins d'amélioration ou d'adaptation à envisager. La parole

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Néanmoins, le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement prévoit une possibilité de régulation de cette espèce dans certains départements, quand les tirs sont possibles.

Aujourd'hui, les comptages annuels démontrent clairement que cet oiseau n'est plus menacé. De plus, selon un rapport produit à la demande du ministre de la transition écologique, les effectifs du cormoran en bord de lac et de

La régulation, par le tir de 290 oiseaux par an, permet toutefois de limiter l'impact nuisible de cette espèce. Cette pullulation est à l'origine de ravages dans les écosystèmes aquatiques et menace désormais les activités piscicoles et l'équilibre de la faune sauvage des zones aquatiques ainsi que la préservation de certaines espèces rares de poissons.

Ce projet de « quota zéro » de prélèvement de cormorans ne va pas dans le sens de la préservation de la biodiversité et pourrait même avoir de graves conséquences sur celle-ci dans mon département. Aussi, je vous demande, madame la ministre, ce que compte faire le Gouvernement pour réguler la population des cormorans et protéger les espèces piscicoles

terres. La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Sido, vous avez interrogé le ministre Christophe Béchu, qui, ne pouvant être présent, m'a chargée de vous répondre. L'arrêté ministériel-cadre du 26 novembre 2010 fixe les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées pour les cormorans. Il est complété par un arrêté pris tous les trois ans fixant les quotas départementaux dans les limites desquels les dérogations peuvent être accordées. À ce jour, quinze arrêtés préfectoraux relatifs aux dérogations sur les cours d'eau et plans d'eau ont été annulés et cinq contentieux sont en attente de jugement. Le groupe national cormorans (GNC) a été chargé de préparer le dernier arrêté triennal, pris le 1 octobre Celui-ci constitue une réponse adéquate aux destructions causées par les grands cormorans sur les cours d'eau et plans d'eau, dans un contexte marqué au cours des dernières années par de nombreux recours contentieux, tous perdus par l'État. Au regard de la difficulté à justifier l'octroi de dérogations sur les cours d'eau et plans d'eau, il a été décidé de proposer un arrêté triennal ne comprenant que des plafonds pour la prévention des dommages pour la pisciculture, sans prévoir de dérogation en dehors de ce secteur. Toutefois, si des études robustes produites localement démontraient l'impact du grand cormoran sur l'état de conservation des espèces

entre 1965 et 1970, des milliers de tonnes de déchets contaminés au lindane provenant de l'usine PCUK de Huningue ont ainsi été accumulées sur le site de la gravière Brunner, au nord de la commune de Sierentz, dans le Haut-Rhin. Si cette entreprise a cessé ses activités depuis cette époque, les inquiétudes concernant une potentielle contamination de la nappe, elles, subsistent. Les dernières vagues de chaleur, l'augmentation de la fréquence de ces dernières et les sécheresses qui les accompagnent n'ont fait qu'accentuer ces inquiétudes au sein de la population et parmi les élus. Ces phénomènes nous rappellent rappellent la rareté et la fragilité de la ressource en eau et l'importance de préserver celle-ci. Si le ministre de la transition écologique a bel et bien décidé d'engager 50 millions d'euros sur cinq pour la dépollution de plusieurs sites contaminés au lindane, celui de Sierentz, lui, ne fait l'objet d'aucune mesure. Parmi les explications avancées pour justifier son exclusion figure le coût de son éventuelle dépollution.

vous avez interrogé le ministre Christophe Béchu, qui me charge de vous répondre en son absence. La gravière de Brunner, située sur la commune de Sierentz, a été comblée dans les années 1960 par les déchets de fabrication du lindane en provenance de l'usine PCUK.

En 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a consacré une enveloppe de 50 millions d'euros sur cinq ans à la poursuite de la reconquête de la qualité de la nappe phréatique d'Alsace. Vous m'interrogez sur l'exclusion de ce site de ce plan d'action. Trois sites prioritaires ont été sélectionnés selon trois critères, parmi lesquels figure, au premier chef, l'impact du site sur la qualité des eaux souterraines. Or la surveillance du site de Sierentz ne montre aucun impact significatif des déchets enfouis sur les eaux souterraines et le coût d'un chantier d'excavation s'élèverait à environ 40 millions d'euros, pour des produits bien moins concentrés qu'à Wintzenheim, par exemple. C'est pour cette raison que le site de Sierentz n'a pu être retenu. Pour autant, l'Ademe accompagne les collectivités, je le rappelle, en finançant la réalisation d'un plan de gestion sur la gravière à proximité du site, dans le cadre d'un projet de renaturation porté par la ville de Sierentz.

la France se dote, depuis plusieurs années, d'un arsenal législatif visant à poser les bases d'un nouveau mode de fonctionnement, plus vertueux, notamment du point de vue de la construction et de la mobilité. Les collectivités territoriales sont pleinement impliquées dans cette transition énergétique et écologique, du fait de leurs compétences, mais également de leur proximité avec les citoyens, qui facilite l'acceptabilité d'une évolution que nous ne devons plus différer. Malgré tout, les élus locaux sont parfois confrontés à des difficultés. C'est notamment le cas avec la rénovation des logements en secteur sauvegardé, qui concerne 46 % des communes. Dans de tels périmètres, les travaux d'isolation, d'installation de panneaux photovoltaïques ou encore la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques peuvent se heurter aux préconisations de sauvegarde du patrimoine.

dans des espaces protégés au titre du code du patrimoine. Toutefois, en séance, cette disposition a été supprimée avec le soutien du Gouvernement. Or les élus locaux craignent que, en raison de contraintes toujours plus exigeantes, les bailleurs publics et privés ne délaissent les centres-villes historiques, alors même qu'ils travaillent assidûment à leur redynamisation. En outre, ces secteurs sont parfois l'atout principal de l'attractivité d'un territoire. Par ailleurs, si les travaux ne sont pas réalisés dans les secteurs sauvegardés, un nombre croissant de bâtiments resteront énergivores et ne trouveront plus preneurs. Or nos quartiers anciens sont en constante évolution depuis des siècles et ils peuvent participer pleinement à cette nouvelle vision de la cité, à la fois durable et vivante. Face à l'importance des enjeux, les acteurs publics et privés doivent pouvoir travailler en bonne intelligence avec les architectes des Bâtiments de France ; de même, les différents documents d'urbanisme doivent faire cohabiter ces deux exigences préserver notre patrimoine bâti ancien et prendre le virage indispensable de la sobriété énergétique. Je souhaiterais donc savoir ce qu'envisage le Gouvernement pour concilier à la fois la protection du patrimoine et l'adaptation de nos villes et villages à la transition écologique. La parole

fait effectivement l'objet de mesures de protection, afin de garantir la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de notre nation. Le Gouvernement a pleinement conscience de la nécessité de concilier concilier la protection du patrimoine et les objectifs de rénovation énergétique et d'élimination des passoires thermiques. Les propriétaires de ces bâtiments patrimoniaux doivent désormais engager des travaux de rénovation énergétique pour conserver la possibilité de mettre en location des logements lorsque ceux-ci sont peu peu performants. Quand il s'agit de locaux tertiaires, ces bâtiments ont des objectifs ambitieux de réduction des consommations d'énergie, dans le cadre du dispositif Éco-énergie tertiaire. La réglementation en vigueur prévoit déjà des mécanismes spécifiques pour tenir compte des contraintes patrimoniales. Néanmoins notre objectif n'est pas d'écarter trop systématiquement les bâtiments patrimoniaux ou historiques de la vague de rénovation. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires travaille donc avec le ministre de la culture pour promouvoir la réalisation de programmes de rénovation énergétique adaptés aux spécificités des bâtiments patrimoniaux. passe, par exemple, par la rédaction d'un guide technique concernant l'implantation de panneaux photovoltaïques en façade ou en toiture, rédigé avec le concours de représentants des architectes des Bâtiments de France, ou par la promotion de techniques de rénovation respectueuses de ces ouvrages, dans le cadre de l'expérimentation du label BBC Effinergie rénovation patrimoine ». Le Gouvernement entend donc contribuer à diffuser les bonnes pratiques et à encourager une rénovation énergétique respectueuse du patrimoine, pour maintenir l'attractivité et le dynamisme de nos centres historiques.

l'objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2050 s'appuie essentiellement sur les collectivités, afin de préserver les espaces naturels et de lutter contre les émissions de dioxyde de carbone. Les acteurs concernés sont tous conscients de l'impérieuse nécessité de modifier nos organisations pour faire face à l'enjeu de la transition écologique. Aussi, aucun d'entre eux ne conteste le but fixé. Toutefois, malgré les avis négatifs du Conseil national d'évaluation des normes,

Les précisions ainsi apportées risquent de léser considérablement les communes rurales, qui doivent pourtant déjà faire face aux enjeux d'accès aux services publics et de lutte contre les déserts médicaux. ailleurs, ce nouveau dispositif changera profondément la façon de concevoir notre aménagement du territoire. Aussi est-il indispensable de proposer des mesures d'accompagnement et de conseil permettant aux maires et aux présidents de nos communautés de communes de se saisir de cette nouvelle façon de concevoir leur développement.

La Première ministre a annoncé plusieurs mesures pour territorialiser et différencier nos objectifs, en clôture du salon des maires, le 24 novembre 2022, à l'issue du travail de concertation mené sous l'égide du ministre Christophe Béchu avec les collectivités et et les parlementaires. Elle s'est notamment engagée à une « prise en compte spécifique des territoires ruraux », la déclinaison territoriale de l'objectif ne devant pas conduire à priver complètement une commune rurale d'une capacité Elle a aussi confirmé que les projets d'envergure nationale seraient comptabilisés non à l'échelle de chaque région, mais bien à l'échelle nationale. Le décret relatif à la nomenclature sera, quant à lui, adapté pour être plus lisible et plus opérant. En cas de blocage à l'échelle d'un territoire, des contrats entre l'État et le bloc communal pourront également être conclus, afin de permettre un équilibre entre développement de projets d'intérêts majeurs et sobriété foncière.

au sujet de l'élargissement des dérogations préfectorales pour les diplômés du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). En effet, en France, lors de l'été 2021, quelque 1 480 noyades accidentelles ont été recensées ; un quart de ces noyades ont entraîné un décès. 47 % ont eu lieu en mer, 26 % en piscine, 23 % en cours d'eau et 4 % dans d'autres lieux domestiques. Ces chiffres, bien qu'en baisse, s'expliquent en grande partie par la reprise des activités sportives en sortie de crise du covid-19, avec des personnes pas toujours réhabituées à l'effort physique. Il est donc crucial d'organiser au mieux la surveillance des baigneurs. Or, en France, nous devons collectivement faire face à une pénurie de maîtres-nageurs ; il en manque 5 000 selon la Fédération française de natation. Certaines piscines sont contraintes de fermer. Plusieurs facteurs expliquent cette pénurie : manque d'attractivité, rémunération peu élevée, mais, surtout, exigences en matière de formation. À l'heure actuelle, il faut disposer d'un brevet d'État d'éducateur sportif aux activités de la natation (BEESAN) ou d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport pour exercer dans un centre aquatique. Toutefois, il est devenu particulièrement difficile de trouver un titulaire de ces diplômes. Ainsi, des dérogations préfectorales ont été mises en place pour permettre aux détenteurs du BNSSA de surveiller les bassins.

associant les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ainsi que les collectivités locales. Ces états généraux permettront d'identifier les évolutions réglementaires que le ministère pourrait entériner à court terme pour résoudre les difficultés d'organisation de la surveillance des activités aquatiques dans les zones de baignade d'accès payant. De plus, ils permettront de définir des axes de promotion du métier de MNS visant à en améliorer rapidement l'image et l'attractivité. Par ailleurs, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'avis favorable émis par le Conseil national d'évaluation des normes relatif à la surveillance, en autonomie, des baignades d'accès payant par les titulaires du BNSSA. Ils visent à dégager des ressources pour l'apprentissage de la natation

Coeur d'Occitanie porté par la chambre de commerce et d'industrie. Il a, depuis, été transmis aux services de la direction générale de l'aviation civile, qui l'ont validé en janvier 2022 comme obligation de service public. reçue aimablement le 12 octobre dernier au cabinet de M. le ministre délégué. Ce dernier devait relancer l'instruction du projet par ses services et ceux de la Commission européenne.

entre Carcassonne et Paris-Orly, et vous demandez quelles mesures l'État entend prendre pour imposer des obligations de service public sur cette liaison. Le règlement européen n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, qui régit le marché libéralisé des services aériens en Europe, permet aux États membres d'introduire des OSP dans

Avant toute publication d'OSP, la Commission surveille le respect des lignes directrices interprétatives du règlement, notamment le caractère vital de la liaison concernée pour le développement économique et social de la région desservie,

la région Occitanie a demandé au ministre de la transition écologique l'édiction d'obligation de service public sur les services aériens réguliers entre Carcassonne et Paris-Orly. La vérification du respect des critères minimaux définis dans le règlement européen et relatifs au caractère vital pour le développement économique et social de la région ainsi qu'à l'absence de moyens de transport alternatifs comparables est en cours ; nous vous l'avons indiqué lors de notre rendez-vous. De premiers compléments d'information ont été apportés en octobre 2021 par la région Occitanie, notamment sur les temps de trajet avec les aéroports proches de Carcassonne desservant déjà la capitale, tels que ceux de Toulouse, de Montpellier, de Perpignan, ou encore de Castres dont la liaison avec Paris est déjà placée sous OSP. La proportionnalité entre la demande de transport estimée et la fréquence souhaitée par les collectivités locales fait l'objet d'études complémentaires. Si une enquête a été lancée au premier trimestre de 2022 par la région Occitanie auprès du tissu économique local pour objectiver le dimensionnement du service, les services de la direction générale de l'aviation civile n'ont pas encore eu communication des résultats de cette étude. La démonstration à faire de cette proportionnalité est importante dans le contexte occitan, dans la mesure où la région compte actuellement trois liaisons d'aménagement du territoire financées par des fonds publics, à savoir les lignes entre Paris-Orly et Rodez, Castres et Tarbes. En outre, l'aéroport de Toulouse, bien que situé à plus d'une heure de route en heure de pointe, propose des vols très fréquents vers Paris, grâce, notamment, à la navette Air France.

chargé des transports. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les nuisances occasionnées par l'aéroport d'Orly, dénoncées tant par les riverains que par les élus locaux du Val-de-Marne et de l'Essonne. La situation de l'aéroport d'Orly est unique en France. Implanté sur une emprise de 1 500 hectares, il est enclavé dans un tissu urbain dense qui préexistait à la construction de cette plateforme. De fait, plus de 2 millions de Franciliens habitent à proximité. Ce statut particulier se traduit par l'existence d'un couvre-feu et d'un plafonnement du trafic aérien désormais garanti par la loi. Or, dans le contexte post-covid-19 du redémarrage de l'économie, le développement d'Orly inquiète, malgré l'adoption le 17 mars 2022 du plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). En effet, le trafic aérien a augmenté de 7 % durant l'été 2022 par rapport à l'été 2019,

de Paris-Orly est plafonné à 250 000 créneaux par an depuis 1994. En ce qui concerne le couvre-feu sur la plateforme de Paris-Orly, il convient de rappeler que les autorités de l'aviation civile veillent à sa stricte application. Toutefois, certains aléas d'exploitation les conduisent à accorder à titre exceptionnel et en nombre très limité des dérogations à son application. Durant les mois d'été, il a effectivement été constaté une augmentation des demandes de dérogation au couvre-feu par rapport à l'année précédente. Celles qui ont été accordées et suivies d'effet l'ont été pour des raisons impératives de sécurité ou des cas de force majeure, comme l'évitement de conditions météorologiques dangereuses ou une urgence médicale, occasionnant des retards à l'arrivée de l'avion. En outre, les mesures inscrites dans le PPBE de l'aérodrome de Paris-Orly le PPBE de l'aérodrome de Paris-Orly pour la période allant de 2018 à 2023 contribuent directement à lutter contre les conséquences sanitaires du bruit aérien. Le PPBE de Paris-Orly contient un objectif de réduction de bruit quantifié : diminuer de six décibels le niveau sonore heures à six heures, et réduire de 50 % les populations exposées à une forte perturbation du sommeil. Pour ce faire, d'éventuelles restrictions d'exploitation pourraient être mises en place en fonction des conclusions de l'étude d'impact qui a été menée, dans une approche équilibrée, réalisée conformément à la réglementation européenne. Cette étude a été engagée en 2019 pour analyser les effets de plusieurs scénarii de restrictions d'exploitation. Alors qu'elle était sur le point d'aboutir, elle a dû être retardée en raison des effets de la crise sanitaire qui ont ralenti les travaux relatifs à l'élaboration du PPBE, dont l'adoption est un préalable indispensable à toute étude d'impact. Dès l'adoption du PPBE, l'étude d'impact permettra de dégager les solutions adaptées à la situation locale, et proportionnées aux enjeux socio-économiques du territoire desservi par l'aéroport.

Depuis la mise en service de la ligne en juillet 2017, les travaux inhérents à la création de la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire sont terminés. Pour ce chantier, SNCF Réseau a acheté de nombreux terrains. Les habitants et les communes concernés devaient avoir la possibilité de racheter ces terrains non utilisés, appelés « excédents d'emprise » ou « délaissés ». L'importance d'un traitement dynamique de ces dossiers de terrains délaissés par la SNCF avait été soulignée à de nombreuses reprises, car ils étaient susceptibles d'être remis à la disposition des collectivités, des entreprises et des administrés. Il est essentiel de rappeler que SNCF Réseau s'est engagé auprès des communes à prendre en charge le bornage et les frais afférents, mais pas uniquement. En effet, dans le cadre des procédures de déclassement des voiries qui jouxtent les terrains vendus, voire les traversent, certaines communes se retrouvent toujours à devoir gérer techniquement et financièrement ces procédures qui ont un coût. Alors que cette charge relève exclusivement du projet mené sur l'initiative de SNCF Réseau et de ses partenaires, dont Eiffage, des solutions concrètes doivent être proposées aux communes démunies et désabusées. J'en appelle au respect des engagements pris. Les Les maires des communes concernées, traversées par la LGV, trouvent le temps long et souhaiteraient que les parcelles achetées à l'époque puissent, enfin, être vendues aux personnes intéressées, comme cela leur avait été annoncé.

SNCF Réseau a dû acquérir pour la construction de cette ligne nouvelle des parcelles dont l'emprise totale, indispensable pour la réalisation des travaux, ne serait pas nécessaire à terme pour l'exploitation de la ligne. Lors de la phase de conception, il avait été effectivement convenu que celles-ci, une fois les travaux terminés, seraient revendues en priorité aux collectivités concernées ou aux habitants et entreprises des communes sur lesquelles elles sont situées. Ces délaissés ferroviaires représentent 1 000 hectares répartis dans cinquante-six communes à l'échelle du projet. Ainsi, dès 2019, SNCF Réseau a entamé des procédures de revente de ces parcelles en tenant compte de contraintes liées aux réserves de foncier nécessaires au parachèvement de la LGV, notamment la mise en oeuvre d'un dispositif exceptionnel de lutte contre les pics de bruit mis en place, à la demande du Gouvernement, pour traiter les situations les plus sensibles. Sa mise en oeuvre a pu, dans certains cas, nécessiter la mobilisation de terrains déjà acquis par SNCF Réseau, et ainsi freiner les reventes de délaissés ferroviaires. Toutefois, à ce jour, les démarches engagées par SNCF Réseau ont significativement progressé : les ventes ou promesses de vente représentent à ce stade 80 % des terrains excédentaires recensés, ces derniers étant systématiquement proposés en priorité aux agriculteurs riverains de la ligne et aux communes concernées. S'agissant des frais de notaires, ceux-ci sont intégrés aux actes administratifs de vente et pris en charge intégralement par SNCF Réseau. Enfin, conformément à ses engagements, lors de chaque revente, SNCF Réseau a fait réaliser le bornage entre le domaine ferroviaire conservé et les parcelles revendues.

régional (TER) reliant Laon à Paris m'ont de nouveau interpellée pour me faire part de leur ras-le-bol face à la dégradation du service : sur le seul mois d'août 2022, ils ont relevé soixante-quatre incidents avec, chaque jour, plus de deux trains connaissant des retards ou des annulations. Cette ligne est révélatrice du calvaire que vivent les 200 000 voyageurs quotidiens des TER des Hauts-de-France, qui supportent des retards et annulations à répétition, mais aussi le manque de place, l'insécurité ou encore une propreté douteuse. Cette situation est le résultat d'un sous-investissement chronique, tant matériel qu'humain. Nos concitoyens vivant en milieu rural sont abandonnés, délaissés. Madame la ministre, notre région semble clairement oubliée des pouvoirs publics. Interrogé au Sénat le 14 septembre dernier, le PDG de la SNCF a lui-même reconnu les défaillances de son déclarant : « On s'est plantés plus lourdement en Hauts-de-France qu'ailleurs. » Xavier Bertrand a annoncé il y a dix jours que la région pourrait de nouveau suspendre ses paiements à la SNCF face à ce trafic dégradé.

Depuis plusieurs mois, les TER des Hauts-de-France connaissent des difficultés de production, entraînant une régularité dégradée ou des trains supprimés. Les problèmes ont notamment trait à l'indisponibilité de rames et de personnels, avec des difficultés de recrutement et des formations retardées pendant la crise sanitaire. Concernant le matériel roulant, SNCF Voyageurs a adapté l'organisation de la maintenance des rames afin de retrouver la disponibilité attendue. Concernant les effectifs, l'entreprise a lancé un plan exceptionnel de recrutement de 440 agents en 2022, dont 110 agents de conduite. plus des trois quarts des recrutements sont couverts. En renfort, des conducteurs d'autres régions et des volontaires récemment partis à la retraite sont sollicités. Néanmoins, il faut être conscient que, la formation durant au minimum un an, le manque de conducteurs ne peut être absorbé que progressivement. Depuis fin octobre, un plan de transport adapté a été mis en place pour sécuriser la circulation des trains les plus fréquentés et réduire le nombre de trains supprimés au dernier moment. Grâce à l'arrivée de nouveaux conducteurs, l'entreprise assure déjà 90 % des trains prévus au plan de transport nominal, et compte résorber progressivement les trains manquants d'ici au troisième trimestre de 2023. Le Gouvernement souhaite que les efforts soient encore intensifiés afin d'envisager une date de retour à la normale anticipée. De surcroît, l'entreprise s'est engagée à communiquer régulièrement les résultats de ce plan de redressement aux associations de voyageurs et aux élus. Je fais confiance à la région Hauts-de-France, compétente pour l'organisation des TER, pour suivre de près ces travaux de la SNCF et répondre aux besoins des habitants de la région. La parole est à Mme Pascale Gruny,

françaises. Franchement, il faudrait plutôt investir dans nos lignes : nos usagers ont tout de même le droit d'aller travailler ! Oui, simplement aller travailler ! Vous parlez de formation et de personnel.

alors même que l'état du réseau ferroviaire rend nécessaire un investissement de 100 milliards d'euros sur quinze ans. Alors que nous n'atteignons pas nos objectifs en matière de report modal ou encore de planification ambitieuse et financée de la politique cyclable, il est temps de réorienter les investissements vers les mobilités utiles et durables.

Toujours en Isère, la création d'un demi-échangeur Vienne Sud sacrifie les habitants de la commune de Reventin-Vaugris alors qu'une alternative réaliste et efficace existe. Autre exemple, en Haute-Loire, l'inutile chantier du contournement de la RN88 détruit les terres agricoles sans la moindre considération. ministre, quelle est votre position sur la demande de moratoire des projets routiers et autoroutiers, et la nécessité de les réexaminer au regard tant des stratégies fixées par l'État que des enjeux climatiques, écologiques et sanitaires auxquels nous faisons face ?

est le sens des nombreuses initiatives lancées en matière de décarbonation des transports routiers ou en faveur d'une évolution des mobilités routières, avec le développement du covoiturage et le partage de la voirie en faveur des modes actifs ou des transports en commun. la route représente 90 % des déplacements de personnes et du transport de marchandises, et reste un élément indispensable à la vie de nos territoires. En outre, la situation de la cinquantaine de projets que vous évoquez est extrêmement variée. En effet, les uns dépendent de collectivités locales, les autres sont en service, encore sont reportés à des horizons lointains et ne sont plus étudiés. Ces différences de situation expliquent la nécessité d'une évaluation propre à chaque projet. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement privilégie une approche pragmatique d'analyse au cas par cas des enjeux des projets. Les différentes évaluations socio-économiques et environnementales soumises au public à l'occasion des déclarations d'utilité publique ou des autorisations environnementales permettent d'objectiver les suites à donner à chacun. chacun. Les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures et la construction des prochains volets routiers des contrats de plan État-région permettront de fait un inventaire global des projets en cours. Un moratoire global ne constitue pas une réponse adaptée au regard des enjeux de ces différents projets et des besoins spécifiques de chaque territoire, autant d'impératifs auxquels je sais le Sénat, comme moi, très attaché.

loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium ».

de Pluneret a été créé en 1997 sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL), qui a été liquidée le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lorient. Les familles ont découvert très tardivement la situation non réglementaire de ce site, et ont lancé différentes procédures auprès du tribunal judiciaire comme du tribunal administratif. Celles-ci n'ont toutefois pas permis de trouver une issue à cette situation. La préfecture du Morbihan est informée de cette situation particulière et s'entretient régulièrement avec le maire de Pluneret à ce sujet. Comme vous le soulignez, la commune de Pluneret peut reprendre la gestion directe de ce site, en application des dispositions de l'article 23 de la loi de 2008 relative à la législation funéraire. Afin d'atténuer les conséquences financières de cette opération sur son budget, la commune peut faire application de la disposition de ce même article qui dispose que « les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation

pour armer les polices municipales en pistolets à impulsion électrique (PIE). La société Taser-Axon dispose d'un monopole sur la fabrication de ces pistolets. En France, elle commercialise trois modèles, de trois générations différentes. L'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale sont autorisés à porter et utiliser ces armes, dites de force intermédiaire à létalité réduite. Par ailleurs, l'article R. 511-28 du même code impose aux forces de police municipale d'utiliser uniquement des pistolets dotés d'un système d'enregistrement vidéo et sonore associé au viseur. au viseur. Les modèles de première et deuxième génération ont été dotés d'une batterie amovible dans laquelle était incorporée une caméra, ce qui permettait de respecter la restriction prévue à ce dernier article. Malheureusement, la nouvelle génération n'a pas été conçue avec ce type d'équipement

de se passer de cette arme de force intermédiaire pourtant de plus en plus essentielle dans l'exercice difficile de leurs missions quotidiennes. Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, si le Gouvernement envisage de réviser cet article du code de la sécurité intérieure pour permettre aux forces de police municipale d'être équipées de façon adaptée.

utilisés par les agents de police municipale soient équipés d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur. Elle renvoyait à des caractéristiques techniques qui ne correspondent plus aux produits commercialisés L'exigence d'une caméra associée au viseur posait également des problèmes opérationnels très concrets, puisque l'agent pouvait, par accident, gêner la captation vidéo en visant. Cette difficulté a été portée à la connaissance du ministère de l'intérieur, qui partage votre avis quant à l'utilité des PIE en tant qu'arme de dissuasion et de défense non létale dans le cadre des missions de la police municipale. Afin d'éviter que les collectivités ne se trouvent dans l'impossibilité de se procurer de nouveaux modèles, le code de la sécurité intérieure a été modifié par un décret du 7 novembre 2022. La nouvelle rédaction donne davantage de souplesse aux collectivités, tout en conservant la garantie de l'enregistrement visuel et sonore des interventions. Désormais, Désormais, l'article R. 511-28 du code de la sécurité intérieure prévoit que les PIE utilisés par les agents de police municipale soient équipés de systèmes de contrôle donnant lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté et qu'il déclenche, au plus tard, lors de la mise sous tension du PIE. Les collectivités ont donc maintenant le choix entre plusieurs possibilités et peuvent continuer d'utiliser les anciens modèles ou acquérir

Le village de Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, a été dévasté. Malgré la force de ce phénomène hors norme et les dégâts considérables, le ministre de l'intérieur a d'emblée annoncé que l'état de catastrophe naturelle ne serait pas reconnu, préfet a ensuite confirmé, le phénomène observé n'entrant pas strictement dans les caractéristiques fixées par le code des assurances. Plus précisément, si certaines rafales ont bien dépassé 215 kilomètres par heure, elles se sont concentrées sur un périmètre physique et temporel limité et non pendant dix minutes ou en rafales. moi, madame la ministre, que cette subtilité peut difficilement être comprise et acceptée par les communes, et encore moins par les sinistrés, dont certains ont vu disparaître en moins de dix minutes le fruit d'années de travail ou d'économies. bénéficier du régime de l'état de catastrophe naturelle, ces derniers ne pourront être indemnisés qu'au regard des garanties prévues dans leur contrat d'assurance, au titre de la garantie tempête, dont nombre de dégâts et dommages sont exclus. Certains sinistrés n'étaient même pas assurés, faute de moyens financiers suffisants. Soyons clairs : la formidable solidarité et les autres dispositifs d'aide ne suffiront pas à effacer les préjudices subis. Cette situation, qui n'est pas isolée, met en évidence l'inadéquation des règles et critères régissant le système de caractérisation des catastrophes naturelles au regard de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes- tornades, sécheresse, inondations, mouvements de terrain ... -dont les conséquences sont de plus en plus lourdes et dont le nombre devrait augmenter de 50 % d'ici à 2050.

la ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ? Comptez-vous accorder le bénéfice de l'état de catastrophe naturelle aux communes sinistrées en octobre dernier

le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu dans le village de Bihucourt quelques heures après ces événements dramatiques afin de témoigner du soutien du Gouvernement aux victimes. Les tornades et, plus largement, l'ensemble des phénomènes venteux violents sont en du régime de la garantie catastrophe naturelle dès lors qu'elles ne sont pas associées à un événement cyclonique. En revanche, les dégâts sur les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités, causés par ces vents violents, sont couverts dans le code des assurances

la garantie tempête permet aux sinistrés d'être indemnisés par leur assureur sans qu'aucune intervention préalable des pouvoirs publics soit nécessaire. L'État mobilise par ailleurs d'autres dispositifs d'aide au profit de certaines catégories de sinistrés, tels que le régime des calamités agricoles pour les agriculteurs ou la dotation de solidarité en faveur des équipements publics non assurables pour les collectivités territoriales. Enfin, sur l'initiative du ministre de l'intérieur, 22 000 euros de crédits de secours d'extrême urgence ont été mobilisés en quelques jours au profit des trente-trois familles de Bihucourt dont les habitations ont été durablement endommagées par la tornade, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins de toute première nécessité.

et des outre-mer. Madame la ministre, en 2008, le commissariat de plein exercice de Noisy-le-Sec a été déclassé en commissariat subdivisionnaire. les effectifs de police nationale de Noisy-le-Sec n'ont cessé de décroître, passant de 150 officiers et sous-officiers à moins de 80 en l'espace d'une quinzaine d'années. Dans le même temps, la population a augmenté, passant de 38 500 habitants en 2008 à 45 000 aujourd'hui. Le territoire continue d'ailleurs de se développer, puisqu'il accueillera prochainement la ligne 11 du métro et le prolongement du tramway T1. de fonctionnaires au commissariat de Noisy-le-Sec peinent à compenser les mutations. De nombreux postes restent vacants, dont plusieurs de commandement. Aujourd'hui, le commissariat peut envoyer à peine 40 agents sur la voie publique, ce qui ne permet pas toujours à Noisy-le-Sec de bénéficier d'une continuité de service, puisqu'il faut compter avec la répartition entre les différentes brigades, mais aussi avec les congés et les arrêts maladie des fonctionnaires de police.

Malgré la politique volontariste de la ville de Noisy-le-Sec, dont je salue le maire et les agents de police municipale pour leur mobilisation sans relâche, les problèmes persistent. Alors qu'elle est elle-même concernée par des difficultés de recrutement, rappelons que la police municipale ne dispose pas des prérogatives

du développement modal à venir et, surtout, parce qu'il s'agit d'une demande des agents de la police nationale, que je salue, et municipale, du maire, des élus, des commerçants et des citoyens, envisagez-vous le retour d'un commissariat de plein exercice à Noisy-le-Sec

de Noisy-le-Sec. La commune continue cependant de bénéficier de la présence d'un commissariat dit « subdivisionnaire ». Cette organisation particulière présente un double avantage : d'une part, elle maintient la qualité du service aux habitants, qui continuent de disposer de l'implantation d'un service de police de proximité dans leur commune, ouvert toute l'année de jour comme de nuit ; d'autre part, elle offre des mutualisations très fortes entre les commissariats concernés, ce qui permet de renforcer les moyens disponibles pour les interventions lorsque la situation l'exige. Je rappellerai aussi que la circonscription de sécurité de proximité de Bobigny-Noisy-le-Sec dispose, hors renforts départementaux, d'un policier pour 455 habitants. Ce chiffre ne révèle pas de sous-dotation. Noisy-le-Sec bénéficie aussi de l'intervention des effectifs de la sous-direction régionale de la police des transports, qui jouera un rôle important dans le plan de sécurisation des sites des prochains jeux Olympiques pour faire face aux flux accrus de voyageurs. Des opérations spécifiques de sécurisation y sont aussi menées régulièrement, notamment dans les cités du Londeau et de Béthisy. Tout ce travail de fond donne des résultats tangibles. Se limiter aux seuls effectifs d'un commissariat pour mesurer les moyens mobilisés pour assurer les missions de sécurité publique aboutirait donc à un malencontreux effet d'optique. Les complémentarités entre les effectifs locaux et ceux du district de Bobigny, du département ou encore de l'agglomération parisienne apportent une meilleure adaptation du nombre de policiers engagés en fonction des situations rencontrées.

Madame la ministre, en raison de l'augmentation du prix de l'électricité et des enjeux liés à la transition écologique, certaines municipalités envisagent, ou pratiquent déjà, l'extinction totale de l'éclairage public. totale de l'éclairage public. Or celui-ci est indispensable à l'exploitation de la voirie ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes. L'extinction totale de l'éclairage public est susceptible de mettre en cause la responsabilité du maire et de la commune. En effet, les juges peuvent soit établir un lien de causalité entre l'absence d'éclairage et le dommage résultant d'un accident soit estimer que le défaut d'éclairage constitue l'élément aggravant d'un accident. D'après la jurisprudence, le défaut ou l'insuffisance d'éclairage public est également susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Il pourrait enfin être reproché au maire un manquement dans l'exercice de son autorité de police ayant conduit à la commission d'infractions. Le cadre légal et réglementaire, qui n'impose pas aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune, ne semble plus adapté. En outre, la réponse du ministère selon laquelle « il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité » n'apporte pas de fondements objectifs susceptibles d'aider les maires et les collectivités dans l'exercice de leurs compétences. Madame la ministre, pouvez-vous préciser les recommandations du ministère de l'intérieur concernant l'extinction de l'éclairage public, afin de protéger les maires et les collectivités face au risque d'engagement de leur responsabilité ?

le cadre législatif, auquel on reproche souvent son excès de précision, n'impose pas d'obligation d'éclairage aux communes, leur évitant ainsi un coût important et une responsabilité accrue. C'est à la commune de déterminer les lieux nécessitant d'être éclairés. La question de l'éclairage public nécessite de concilier trois objectifs : la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité et, enfin, la nécessaire réduction des consommations d'énergie. En l'absence de prescription législative et réglementaire, le juge administratif admet que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités. Toutefois, en cas de défaut d'éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si, outre la responsabilité du gestionnaire de la voirie, des circonstances particulières témoignant d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Aussi, nonobstant l'arrêté municipal édictant les modalités de mise en oeuvre de l'extinction de l'éclairage public, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visibles de nuit, tels que des panneaux réfléchissants ou clignotants avertissant des dangers. Enfin, la modernisation de l'éclairage public s'accompagne d'une baisse de la facture d'électricité, ce qui permet aux communes de dégager de nouvelles marges de manoeuvre pour cibler les lieux où l'éclairage serait rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. La parole

Des témoignages de plus en plus nombreux nous parviennent quant à l'augmentation du temps d'attente pour disposer d'un rendez-vous en mairie afin d'obtenir un titre d'identité. Ces lenteurs contraignent les Français à des déplacements parfois importants et coûteux pour obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables. Les collectivités territoriales semblent ne pas bénéficier des moyens nécessaires pour suppléer aux fortes démarches. Un administré m'a expliqué avoir dû parcourir plus de cinquante kilomètres pour demander un passeport, qui lui permettra de passer les fêtes de fin d'année dans sa famille à l'étranger. Il n'est pourtant pas certain de disposer de son titre avant la mi-décembre. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'indiquer comment le Gouvernement compte résorber ces délais d'instruction anormalement longs, qui pénalisent les Français, et de m'expliquer les raisons de ces blocages, depuis le rendez-vous en mairie jusqu'à la remise du titre. La parole

pour freiner l'augmentation des délais en matière de délivrance des titres d'identité et de voyage, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a décidé de mettre en place un plan d'urgence en 2022. Des actions sont également conduites pour prévenir une nouvelle crise en 2023. une nouvelle crise en 2023. Le Gouvernement a ainsi pris différentes mesures. Je pense tout d'abord au déploiement d'un moteur national de recherche de rendez-vous permettant aux usagers de connaître les disponibilités sur une zone géographique donnée et de réduire le nombre de rendez-vous non honorés. ensuite à l'incitation à l'enregistrement d'une prédemande en ligne pour limiter la durée des rendez-vous de recueil et augmenter le nombre de rendez-vous assurés. Le Gouvernement a également prévu l'installation, en 2022, de 401 dispositifs de recueil et un plan d'installation de 500 nouveaux dispositifs en 2023.

décidé une augmentation temporaire de l'effectif des services d'instruction de 42 % pour 2022 ; le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et des outre-mer prévoit d'y affecter des effectifs supplémentaires pérennes. la revalorisation exceptionnelle de la dotation « titres sécurisés » à hauteur de 21 millions d'euros à compter de 2023. Vous le voyez, toutes les mesures sont prises pour répondre le mieux possible à cette situation et résorber les retards constatés.

en toute impunité, au niveau non seulement religieux, mais également politique, éducatif et social, ainsi qu'à l'hôpital public. Il n'est pas inutile de rappeler que les Frères musulmans, qui seraient 55 000 sur le territoire français, sont considérés comme une organisation terroriste en Égypte, pays qui a vu naître ce mouvement.

en entrant dans la vie publique, voire politique. [ ...] Ils désirent clairement prendre le pouvoir par les urnes. [ ...] Le but est de faire un jour que le pays dans lequel ils se trouvent soit régi par la loi de Dieu et non par la loi des hommes.

humaines (IESH) de Château-Chinon, censé former des imams et des cadres religieux, est considéré par beaucoup comme la base arrière des Frères musulmans en France. Dans ce contexte préoccupant pour notre sécurité, je m'étonne du mystère autour de la composition du Forum de l'islam de France (Forif) mis en place par le Gouvernement. Je me demande notamment pourquoi la liste de ses membres n'est pas divulguée, mais je me demande surtout si les Frères musulmans en sont bien exclus ! Madame la ministre, quels sont les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour lutter contre cette organisation prosélyte, qui s'inscrit dans le temps long pour parvenir à ses fins ?

la lutte contre le séparatisme islamiste, qu'il soit lié à la mouvance des Frères musulmans ou à d'autres branches, comme le salafisme, est une priorité du Gouvernement. En témoignent les quatorze prédicateurs évoluant dans la mouvance des Frères musulmans qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, tandis que six autres se sont vu refuser le droit d'entrer sur le territoire français. Par ailleurs, depuis 2017, cinq associations évoluant dans la mouvance des Frères musulmans ont été dissoutes. Si nous sommes sans concession avec ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République, nous souhaitons entretenir le dialogue avec nos compatriotes musulmans indépendants et constructifs. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Forum de l'islam de France, que vous que vous avez cité. Cela va dans le sens de la réforme des modalités de dialogue entre l'État et le culte musulman engagée depuis 2003. Les participants au Forif sont des acteurs du culte musulman, ... Lesquels ? ... actifs dans leur territoire, ayant donné leur accord pour travailler au niveau national avec l'État. Le Forif n'est pas une organisation il n'a pas vocation à représenter les musulmans. Il s'agit du regroupement de personnes identifiées par les préfets et engagées pour travailler avec l'État. C'est précisément parce que nous ne désirons pas reproduire les erreurs du passé,

L'objectif est de faire avancer des projets portés par des acteurs de terrain et de faciliter la structuration d'un islam de France émancipé des ingérences étrangères et de l'influence des porteurs de haine.

Dans ce document, la Cour des comptes constate tout d'abord des avancées importantes dont la création d'une agence régionale de santé et d'un rectorat de plein exercice, la relance de la lutte contre l'immigration clandestine, le renforcement des moyens consacrés à la sécurité ou encore la création d'un établissement public foncier et d'aménagement. La Cour des comptes souligne cependant que, malgré ces avancées et un réel rattrapage du niveau de vie des Mahorais, les services de l'État et du département ne parviennent pas à apporter les solutions attendues par les habitants sur le plan social, économique et sociétal. Je souhaiterais savoir, madame la ministre, quelles suites le Gouvernement entend donner aux treize recommandations formulées par la Cour des comptes afin notamment de consolider l'action des pouvoirs publics et de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine

je peux vous affirmer que le Gouvernement est très attentif à la prise en compte des recommandations formulées. S'agissant du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, la stratégie repose, depuis 2019, sur le plan Shikandra 2.0, partenariat civilo-militaire agissant notamment sur la prévention, l'éloignement, la lutte contre la fraude. L'État mobilise des moyens opérationnels renforcés et inédits au plan national. À titre d'exemple, trois intercepteurs sont en permanence en mer et un en alerte. Près de 24 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière l'an passé à Mayotte, soit 78 % de plus qu'en 2020. Je rappelle que la meilleure façon de lutter contre l'immigration clandestine, c'est aussi de favoriser le développement des Comores.

que le port de Longoni est un port départemental et que l'État sera toujours présent pour accompagner, en lien étroit avec le département, le développement de cette infrastructure stratégique pour le territoire. Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que nous sommes attentifs au développement régional de votre territoire, parce que c'est dans ce contexte

ma question porte sur les difficultés que rencontrent les communes rurales à obtenir des propriétaires défaillants d'immeubles identifiés comme dangereux le remboursement des frais qu'elles doivent engager pour faire cesser le péril. En l'espèce, le maire de la commune de Bonson, dans les Alpes-Maritimes, touchée par la déferlante de la tempête Alex en octobre 2020, avait été alerté sur l'état préoccupant d'un bâtiment privé à l'abandon, situé en coeur de village et fortement fragilisé par l'événement. Face à cette situation, le maire diligentait en urgence une entreprise spécialisée, qui concluait à la dangerosité du bâtiment et en avertissait le propriétaire, une société civile immobilière domiciliée à Monaco, qui n'a donné aucune suite, malgré les relances de la mairie. Dès lors, la commune saisissait le tribunal administratif, qui concluait à un péril grave imminent, en même temps qu'il entérinait le relogement anticipé d'une des propriétaires mitoyennes du bâtiment.

y compris à la proposition d'achat du bien qui lui a été faite. Dans le cas d'espèce, Bonson ne peut prétendre à aucune subvention. Une telle situation n'est pas acceptable, moralement et financièrement. Aussi, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette problématique particulière, malheureusement courante dans les villages, et les évolutions qu'il pourrait entreprendre en faveur des communes rurales qui y sont confrontées et qui ont grand besoin d'accompagnement et de soutien,

le Gouvernement est fortement engagé dans la lutte contre l'habitat indigne aux côtés des collectivités. Une ordonnance de 2020 a ainsi refondu le cadre juridique, unifiant plus d'une dizaine de procédures de police administrative utilisées en matière de lutte contre l'habitat indigne, dont la police du péril. Cette nouvelle police permet d'intervenir plus rapidement et plus efficacement sur les situations d'habitat indigne. À ce titre, le maire peut saisir le tribunal administratif pour obtenir la nomination d'un expert dépêché sur place pour dresser la liste des désordres et des mesures nécessaires pour y remédier. Sur le plan financier, les communes bénéficient d'un soutien fort de la part de l'Agence nationale de l'habitat, qui finance 50 % du montant des travaux d'office exécutés sur le fondement d'un arrêté de mise en sécurité. Ce taux est majoré à 100 % sur six départements dits « territoires d'accélérations », dont le département des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il existe différents dispositifs permettant aux communes d'acquérir des logements indignes dans des conditions facilitées. de l'expropriation simplifiée pour les logements frappés d'un arrêté de mise en sécurité comportant une prescription d'interdiction définitive d'habiter ou de démolition. l'espèce, la commune de Bonson peut étudier l'opportunité de lancer une procédure ordinaire de mise en sécurité comportant une interdiction définitive d'habiter, afin d'engager ensuite une expropriation

E en 2034. En 2022, les circonstances ont bien changé : le secteur du bâtiment est confronté à une pénurie de matériaux, les soubresauts du covid-19 ont encore ralenti des décisions d'assemblée générale indispensables pour prévoir des travaux de rénovation énergétique efficaces, et le coût des travaux énergétiques, déjà chers initialement, est décuplé par l'inflation, au moment où la situation du marché du crédit se tend. MaPrimeRénov'est le seul dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Il est aujourd'hui manifeste que, malgré son succès, son succès, cet outil n'accompagne pas efficacement la sortie du statut de passoire énergétique, 2 500 logements seulement étant sortis de ce statut en 2021 ! Depuis juillet 2022, nous savons que 2 millions de logements sont concernés par cette future interdiction de location dans le parc locatif, dont 1,6 million de logements dans le parc privé. Les professionnels de l'immobilier alertent : ils constatent une tension accrue de l'offre locative, à la fois en raison d'une moindre mobilité dans le parc, et de ventes de biens classés F et G à la hausse. Ils estiment à un quart le nombre de logements classés F et G actuellement loués qui seront vendus. Ils alertent en particulier sur le risque observé dans les immeubles, avec des copropriétaires bailleurs qui déplorent de ne pas parvenir à obtenir un vote en assemblée générale de copropriété permettant des travaux de rénovation efficaces, notamment l'isolation par l'extérieur. Les deux tiers des logements très énergivores du parc privé locatif sont situés en copropriété. Ne faut-il pas envisager très vite une stratégie de rénovation pour le parc collectif intégrant la spécificité et le rythme de la copropriété ? En d'autres termes, comment comptez-vous éviter l'écrasement de l'offre locative ? Je vous remercie, ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, le Gouvernement partage l'idée que la rénovation énergétique des copropriétés fait face à un certain nombre de freins dans la prise de décision des travaux et leur réalisation. Ceux-ci sont accentués dans un contexte inflationniste et de hausse des coûts des matériaux. Des aides financières ciblées existent déjà. En 2021, 11 892 logements ont bénéficié du dispositif bénéficié du dispositif MaPrimeRénov'Copropriétés, attribuée par l'Anah pour des travaux de rénovation énergétique. On constate que 27 % de ces logements atteignent une étiquette B, et 11 % des logements sortent du statut de passoire énergétique F ou G. Au début du mois de novembre 2022, quelque 10 270 logements ont bénéficié de MaPrimeRénov' Copropriétés depuis le début de l'année, ce qui signifie que le dispositif sera en progression cette année. Les moyens consacrés par l'Anah à ce dispositif seront augmentés en 2023 et, en complément, il est possible de mobiliser des CEE d'économie d'énergie), ou le prêt éco-PTZ copropriétés. L'accélération de la rénovation des copropriétés est une priorité pour les prochaines années. En complémentarité des aides financières, il est nécessaire de mettre à disposition un accompagnement structuré autour du service public de la rénovation France Rénov'et des filières professionnelles, notamment les syndics de copropriétés. Il faut aussi réfléchir à la gouvernance des copropriétés, qui peut conduire à des blocages. Une mission sera confiée à l'inspection générale du développement durable (IGEDD), afin d'identifier les freins actuels à la rénovation énergétique des copropriétés et faire des propositions de voies d'amélioration.

Ni la loi Climat et résilience, ni les textes budgétaires qui ont suivi, ni encore moins les décrets d'application pris à la hâte par le Gouvernement et faisant l'objet d'un grave contentieux ne donnent aux collectivités locales une vision claire sur les outils et les moyens d'y parvenir, alors même que l'impact pour les collectivités s'annonce majeur. Leurs ressources et leurs modes de financement actuels ne sont absolument pas adaptés à l'atteinte de cet objectif. La définition d'un modèle économique s'avère ainsi d'une impérieuse et urgente nécessité. En effet, la suppression de la taxe d'habitation ou encore les injonctions contradictoires de l'État incitant, d'un côté, les communes à accroître leur stock de logements sociaux et, d'un autre côté, à réduire leur consommation de foncier, ne font que fragiliser leurs finances. La pression foncière joue en défaveur des terres naturelles et agricoles et il est moins coûteux de construire des logements neufs éloignés des centres-villes que de reconstruire « la ville sur la ville Comme trop souvent, l'État se borne à adresser de grandes injonctions aux collectivités, sans considérer les impacts pratiques et locaux. Avec un financement des communes en grande partie artificialisant, puisque fondé sur le foncier et le développement urbain - rappelons que sur les 230 milliards d'euros collectés au titre de la fiscalité locale, les deux tiers reposent sur le foncier -, l'application du ZAN enrayera la dynamique économique des collectivités locales. C'est tout un modèle économique qui est ici remis en question et toute une politique fiscale qu'il faut revoir. Après l'excellent rapport rendu par mon collègue Jean-Baptiste Blanc sur ce sujet, je souhaiterais donc savoir par quels leviers économiques et fiscaux

Les conséquences sont écologiques, mais aussi socioéconomiques. La France s'est donc fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette » des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années, à l'horizon de 2030. Pour accompagner les territoires engagés vers la sobriété foncière,

le remettre en état et le porter avant revente à une collectivité, en mobilisant les recettes de la taxe spéciale d'équipement (TSE). Des aménagements des dispositifs fiscaux ont par ailleurs été mis en oeuvre pour inciter à une plus grande sobriété foncière : abattement : abattement de plus-value immobilière pour les opérations de surélévation, ainsi que les opérations de recyclage urbain dans des secteurs de contrats entre l'État et les collectivités. Mais il faut sans doute aller plus loin, notamment en s'appuyant sur les travaux du Parlement, en lien étroit avec les collectivités territoriales. Je l'ai indiqué en répondant à la question du sénateur Vaugrenard, le Gouvernement travaille

leur centrale. Celles-ci doivent gérer l'afflux de population et de travailleurs par la construction et la gestion de bâtiments et infrastructures publiques adaptés, être en mesure de supporter dans des conditions de sécurité maximale les flux routiers, le stationnement, et assurer au mieux la gestion des risques. L'ensemble de ces missions nécessite des moyens en termes d'ingénierie, de ressources humaines et de temps de mobilisation des élus, parfois dans des communes de faible importance. Par ailleurs, les dispositions de la loi NOTRe prévoient le surclassement des communes touristiques, stations balnéaires classées et des communes dotées de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ce qui donne aux élus les moyens de conduire une politique de développement local plus adaptée. adaptée. Donner la possibilité d'un surclassement aux communes sièges d'un centre nucléaire de production d'électricité leur donnerait accès à des moyens auxquels elles aspirent pour une meilleure gestion de leur collectivité, tels que le recrutement d'un directeur général des services plutôt que d'un secrétaire de mairie,

de taille comparable. Le Gouvernement envisage-t-il de permettre aux communes hébergeant un centre nucléaire de production d'électricité de bénéficier d'un classement dans une strate de population supérieure à celle enregistrée par l'Insee ?

: si les communes sont classées stations de tourisme ou si elles comprennent sur leur territoire au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. L'objectif du législateur dans ces deux cas est bien de permettre aux communes de faire face à des contraintes particulières, pérennes ou temporaires. Le surclassement démographique leur permet de bénéficier de moyens supplémentaires et, notamment, de créer des emplois fonctionnels supérieurs à ce qu'autoriserait leur strate démographique. Il ouvre aussi droit à une majoration des indemnités des élus locaux. En revanche, le surclassement ne conduit à aucune dotation supplémentaire de la part de l'État. À cet égard, faire bénéficier d'un surclassement démographique les communes accueillant sur leur territoire une centrale nucléaire s'écarte sensiblement des motifs qui justifient ce dispositif dérogatoire. De plus, la sécurité nucléaire étant une question régalienne qui reste du ressort du Gouvernement, les contraintes liées à la présence d'une centrale nucléaire ne semblent pas de nature à faire peser une charge disproportionnée sur la commune. Ces contraintes, si tant est qu'elles soient avérées, ne sauraient en tout état de cause trouver une réponse adaptée dans un surclassement démographique. Vous conviendrez enfin avec moi, monsieur le sénateur, que la présence d'une centrale nucléaire est aussi une source de développement. Un établissement de cette nature emploie un personnel permanent et qualifié, dont la présence est favorable à l'économie locale et contribue aux recettes fiscales des collectivités.

Cet aéroport important pour le tissu économique de la métropole européenne de Lille, du département du Nord et de la région Hauts-de-France fait l'objet d'un projet de modernisation permettant notamment la mise aux normes européennes de sécurité, l'amélioration de l'accueil des passagers, ainsi que l'augmentation de la fréquentation, qui passera de 2,2 millions de passagers en 2019 à 3,9 millions en 2039, occasionnant ainsi plus de 4 000 mouvements supplémentaires par an. Toutefois, les nuisances sonores que subissent déjà les riverains des communes du sud de la métropole du fait de l'activité de l'aéroport

Dans l'optique d'allier la réduction des nuisances au développement de l'aéroport, il me semble de bon aloi de prendre une décision ministérielle interdisant l'utilisation de nuit, entre vingt-trois heures et en application de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, sur le modèle de la décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly.

vous me demandez l'application d'un couvre-feu sur la plateforme pour réduire les nuisances sonores engendrées par son activité, tout en maintenant les conditions de son développement. Cet aéroport décentralisé, quinzième de France par le nombre de mouvements commerciaux en 2021, fait l'objet d'un projet de mise en conformité aux normes de sécurité et de sûreté et d'amélioration des conditions d'accueil des passagers, qui sont en nombre croissant. Ce projet est source d'inquiétude pour les populations riveraines, en particulier du fait des nuisances sonores et environnementales qui en découleraient. Les attentes qui ont été exprimées par les habitants comme par les élus du territoire, notamment dans le cadre de l'enquête publique, sont très fortes. Je les ai entendues et c'est pourquoi le Gouvernement a souhaité y répondre. La ministre chargée des transports a ainsi demandé à ses services que commence sans tarder l'étude visant à évaluer l'efficacité et la proportionnalité de la mise en place de mesures de réduction du bruit et d'éventuelles nouvelles restrictions d'exploitation sur l'aéroport de Lille-Lesquin. Il s'agit d'une étude d'impact prévue par la réglementation, et c'est le préfet du Nord qui la pilotera. Elle comportera une phase de consultations à laquelle toutes les parties prenantes du territoire seront associées. Elle permettra de déterminer, en concertation, des mesures de réduction des nuisances et de protection de l'environnement équilibrées, c'est-à-dire adaptées à l'environnement de l'aéroport et proportionnées au regard des besoins socioéconomiques du territoire desservi.

l'heure où les professions de santé font face à des difficultés majeures, le corps des sages-femmes se retrouve fragilisé et divisé au sein même de la fonction publique. Celles et ceux qui exercent dans les centres de planification et d'éducation familiale et les centres de PMI ne perçoivent toujours pas la prime de complément de traitement indiciaire de 183 euros mensuels, et restent dans l'attente de l'application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022. En revanche, les sages-femmes hospitalières en bénéficient depuis plus de deux ans De plus, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le bénéfice de la prime d'exercice médical de 240 euros mensuels aux sages-femmes territoriales, leur mission n'étant pas assimilable à celle des sages-femmes Elles exercent pourtant le même travail, avec le même diplôme. Elles ne pratiquent pas, certes, les accouchements, mais assurent le suivi obstétrique et gynécologique auprès d'un public fragile. pallient également la crise de l'hôpital sur certains territoires en tension. Cette disparité au sein de la profession nourrit un sentiment de dévalorisation pour ces soignants, qui assument les mêmes responsabilités médicales dans l'accompagnement de nos concitoyennes. Une telle situation pénalise des professionnels qui ont choisi le service public de santé pour tous. Il s'agit de garantir aux sages-femmes, quels que soient leur statut et leur lieu d'exercice, la reconnaissance qu'elles méritent. Pourquoi, madame la ministre, attendre pour rétablir l'équité au sein du métier ?

ne pouvant être présent, m'a chargée de vous répondre. Le Gouvernement s'est pleinement engagé depuis la signature des accords du Ségur de la santé à mieux reconnaître les compétences

C'est ainsi qu'un protocole d'accord signé le 22 novembre 2021 prévoit une revalorisation des grilles indiciaires des sages-femmes hospitalières. Cette revalorisation s'applique également, depuis avril 2022, aux sages-femmes territoriales, de manière obligatoire, et indépendamment de l'établissement ou du service dans lequel elles travaillent. Il n'est cependant pas prévu d'étendre aux sages-femmes territoriales le bénéfice de la prime d'exercice médical instaurée dans ce protocole pour les sages-femmes hospitalières. En effet, cette prime vise à reconnaître la spécificité du travail au sein des établissements de santé et à accompagner la création d'une filière médicale. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer à la fonction publique territoriale. En revanche, le complément de traitement indiciaire, qui a été octroyé aux sages-femmes hospitalières, a été étendu aux sages-femmes territoriales par la loi de finances rectificative pour 2022 votée cet été. En conséquence, la majorité des sages-femmes territoriales, par exemple celles qui travaillent dans les services départementaux

Le décret correspondant est en cours de publication. Il s'agit là encore d'un engagement politique fort du Gouvernement, pour revaloriser les métiers du secteur social et médico-social, qui jouent un rôle primordial dans l'accompagnement quotidien des personnes concernées.

défendu cet accompagnement. L'engagement du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse porte sur trois avancées majeures visant à améliorer la situation des AESH et, donc, à créer l'attractivité nécessaire pour recruter, mais aussi pour fidéliser

Centenaires pour certains, les jardins d'enfants ont bénéficié d'une dérogation à l'obligation d'instruction jusqu'à la rentrée de septembre 2023. Ces structures ne peuvent donc plus prendre d'inscriptions pour la rentrée prochaine, laissant beaucoup de familles dans l'incertitude. À Paris, les jardins pédagogiques municipaux sont de vrais vecteurs de mixité sociale. Situés en très grande majorité en quartier populaire, hébergés par les bailleurs sociaux, ils accueillent toutes les familles, quels que soient leurs revenus, celles qui déclarent des revenus inférieurs à 1 000 euros représentant parfois jusqu'à deux tiers des enfants inscrits. également un modèle d'inclusion, puisque les enfants en situation de handicap représentent 13 % des enfants accueillis dans les jardins d'enfants parisiens, soit plus du double de la proportion constatée dans les écoles maternelles. Cet été, le ministre de l'éducation nationale disait vouloir « trouver une solution juridique pour que les jardins d'enfants puissent continuer leur activité et qu'il [ ...] fallait trouver un chemin pour que cela soit soutenable

l'enfant doit être scolarisé ou peut bénéficier, après autorisation, de l'instruction dans la famille. Afin de permettre aux jardins d'enfants, qui accueillent des enfants entre 2 ans et 6 ans, de se transformer, une période transitoire de cinq années leur a été accordée. Cette période prend fin à la rentrée scolaire 2024.

Strasbourg qui compte 775 enfants accueillis dans ces structures. Je tiens à rappeler que l'abaissement de l'âge de l'instruction à 3 ans consacre le modèle de l'école maternelle française, qui est mondialement reconnue par la qualité de l'instruction qu'elle dispense, de sa gratuité, mais aussi de son accessibilité sur l'ensemble du territoire français. Elle permet ainsi à de jeunes élèves de se préparer, dans des conditions

Je constate d'ailleurs qu'à Strasbourg cette transformation est en cours et que l'ensemble des jardins d'enfants deviendront, pour la plupart d'entre eux, des crèches qui accueillent des enfants de 0 à 3 ans ou encore des écoles hors contrat.

Les membres de la commission de la culture du Sénat ont tour à tour exprimé hier, dans l'hémicycle, lors de l'examen des crédits de la mission « Culture » leur profonde inquiétude si des annulations et des reports de festivals se confirmaient en 2024 à cause de l'organisation des jeux Olympiques. Je suis également étonné par la radicalité des déclarations du ministre de l'intérieur, qui nous oblige en définitive à faire le choix entre nos fêtes. Une fois de plus après la polémique de la circulaire Collomb, la culture paye dans tous les sens du terme pour des questions de sécurité, sauf qu'en l'espèce ce n'est pas pour la sienne

La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est explosive. Vous avez réussi à opposer l'Île-de-France aux autres territoires et le sport à la culture ! Le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles dénonce un acte d'« anti-décentralisation » inacceptable. Le Sénat parlerait, sans doute, d'« hypercentralisation Cette verticalité, source de tensions et de fractures au sein de la population, n'est plus acceptable. J'en viens donc à ma question. Se rappelant opportunément les vertus de la concertation,

de lourds moyens techniques. Nos plus importantes manifestations culturelles, en particulier les festivals, sont aujourd'hui sécurisées par le ministère de l'intérieur, car ce sont souvent des événements rassemblant plusieurs milliers de personnes. Il s'agit donc de concilier la vitalité culturelle qui définit la France et l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, qui impliqueront une forte mobilisation en matière de sécurité. C'est le travail que mène actuellement le Gouvernement. La ministre La ministre de la culture a réuni récemment les plus importants organisateurs de festivals et les syndicats d'employeurs pour évoquer l'ensemble des sujets : mobilisation des forces de l'ordre, des bénévoles, tension sur la disponibilité des techniciens et des moyens techniques, transport des festivaliers, etc. Un travail

En vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, lorsqu'une découverte de vestiges archéologiques est faite sur un chantier de construction, des fouilles sont réalisées et assurées par l'aménageur du projet. projet. Certaines de nos communes rencontrent des difficultés dans la prise en charge des fouilles induites par la construction de certains bâtiments. C'est le cas d'Entrammes, en Mayenne, reconnue pour son histoire riche et sa position stratégique. Elle fait donc l'objet d'un suivi particulier par les services d'archéologie.

Les élus de la commune se voient ainsi confrontés à de nombreuses difficultés à la fois en termes de coûts, de délais de moyens et d'opportunités. Il convient de rappeler que la durée de la réalisation d'une telle opération ne peut être réglementée, car elle dépend d'un certain nombre de critères tels que la localisation, la nature des vestiges, la nature des sols,

et social. C'est justement cet équilibre que les élus d'Entrammes souhaitent atteindre. Ils attendent ainsi que les contraintes puissent être limitées, voire amoindries, car ils s'inquiètent de ne plus être en mesure de concilier leur riche passé et le besoin de développement de la commune sans mettre en péril leurs budgets : l'attractivité de leur commune est en jeu

-ou garantissant la préservation du patrimoine. Ces prescriptions s'appuient sur les avis des commissions territoriales de la recherche archéologique afin de garantir que les obligations faites aux aménageurs

L'archéologie préventive dispose donc d'un cadre législatif, réglementaire et financier adapté. Ce dispositif équilibré participe au développement de la politique culturelle, patrimoniale et scientifique soutenue par le ministère de la culture, tout en garantissant un aménagement raisonné du territoire, notamment en milieu rural.

du plan d'investissement France 2030, des mesures qui permettront d'augmenter la production de granulés et a lancé un appel à projets « biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire » (BCIAT). Comment le Gouvernement entend-il amortir l'éventuelle rupture d'approvisionnement

chaufferies liées à la fabrication de granulés pour une puissance de 148 mégawatts, ce qui représente une production annuelle de granulés

Il convient, bien sûr, d'exclure les projets surdimensionnés inadaptés qui transforment nos agriculteurs en énergéticiens au détriment de leur activité première et de notre souveraineté alimentaire.

à la construction de deux hangars photovoltaïques. Leur projet est malheureusement à l'arrêt à la suite d'un arrêté de prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive.

Lors du 104 congrès des maires, la Première ministre s'est engagée à améliorer les zones de revitalisation rurales. La nouvelle ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Mme Dominique Faure, prépare dans ce contexte un second souffle pour l'agenda rural. Une mission

L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence accordé à un conseiller régional pour participer aux séances plénières, aux réunions de commissions ou aux réunions d'organismes où il est désigné pour représenter la région est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effectives pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne seraient pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'État. Je souhaite donc connaître la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional qui utilisent les autorisations d'absence prévues aux articles L. 4135-1 et L. ainsi que les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en oeuvre concrète de cette règle. Cette question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental. La parole est à Mme la

Le Gouvernement est attentif à la bonne application des garanties particulières apportées aux élus locaux pour leur permettre de cumuler l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Le code général des collectivités territoriales prévoit plusieurs dispositifs permettant à ces élus de concilier activité et mandat sans être pénalisés dans l'acquisition des droits et garanties qui en découlent. Les élus locaux bénéficient notamment de deux types de facilités : d'une part, les autorisations d'absence visées aux articles L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers régionaux et L. 3123-1 pour les et L. 3123-1 pour les conseillers départementaux ; d'autre part, les crédits d'heures sont consacrés à l'article L. 4135-2 pour les conseillers régionaux et à l'article L. 3123-2 pour les conseillers départementaux. absences qui résultent de l'utilisation de ces crédits d'heures et autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté et du droit aux prestations sociales. Concernant les droits à pension de retraite des fonctionnaires, ces temps d'absence accordés aux élus locaux doivent donc être reconnus comme du temps passé dans une position statutaire comportant l'accomplissement de services effectifs. Ces temps d'absence doivent donc être pris en compte

Sollicitée par l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales (Adapei) du Doubs, je souhaite vous interroger, madame la ministre, sur les complications quotidiennes que vivent certains de nos concitoyens non-voyants ou malvoyants. Le problème concerne le remplacement progressif des terminaux de paiement électronique (TPE) de carte bleue dont le clavier est doté de touches physiques par des écrans tactiles tels que nous les utilisons sur nos smartphones pour effectuer les règlements par carte bancaire. La digitalisation des pratiques, phénomène accentué par la crise sanitaire liée au covid-19, s'avère inadaptée pour les personnes déficientes visuelles. En l'absence de repères tactiles, il devient impossible pour elles de taper en toute confiance leur code confidentiel. Cette situation conduit bon nombre d'entre elles à devenir dépendantes d'une tierce personne : certaines ont déjà été contraintes de révéler leur code secret aux vendeurs eux-mêmes, ce qui est- vous en conviendrez -inacceptable. Pour cette partie de la population, la démocratisation digitale est non pas signe de progrès, mais synonyme d'exclusion et de marginalisation. Dans ce contexte, de simples achats quotidiens créent un sentiment de vulnérabilité. Aussi, je souhaite savoir quels sont les leviers possibles pour agir de manière concrète sur les conséquences de cette mutation sociétale. Plus précisément, madame la ministre

qui constitue l'une des conditions d'une société inclusive, représente une préoccupation majeure du Gouvernement. Dans cette perspective, le Gouvernement s'est engagé à transposer en droit national, avant la fin de l'année 2022, la directive européenne du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, qui va créer un corpus de règles nouvelles auquel seront assujettis le secteur culturel, celui des transports, mais également le secteur bancaire. Les travaux de transposition vous seront prochainement présentés dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue). Dans ce cadre, les établissements bancaires auront l'obligation d'adapter une large partie des produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs en matière de crédit, de services de paiement, de services d'investissement ou de monnaie électronique, afin que ces derniers soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Ainsi, ces biens et services devront respecter un ensemble de critères tenant compte de la diversité des formes existantes de handicap, et devront garantir leur compatibilité avec les dispositifs d'assistance. Le champ d'application de la directive incluant les terminaux de paiement, le parc de ces terminaux, constitué à ce jour d'environ 1,5 million d'équipements de proximité, fera l'objet de nombreuses évolutions à moyen terme afin de s'adapter à ces obligations nouvelles. Ces évolutions permettront, par ailleurs, d'amplifier la démarche qui avait été engagée dès dès 2019 par les acteurs de la chaîne des paiements afin d'encourager le développement et l'implémentation de TPE accessibles aux personnes en situation de déficience visuelle ou, plus récemment, au travers de la formalisation d'une charte pour l'inclusion dans les paiements. L'accessibilité universelle est l'un des axes principaux de nos travaux préparatoires à la Conférence nationale du handicap qui nous réunira en 2023.

Relais ! », lieu d'accueil, de répit et de loisirs destiné aux enfants porteurs de handicap âgés de 3 ans à 17 ans qui est implanté à Charleville-Mézières, ville chef-lieu des Ardennes, avec un rayonnement sur l'ensemble du département. Ce dispositif a été créé en mai 2020 sur l'initiative de l'association

au confinement. Ce centre, qui peut accueillir simultanément jusqu'à 8 enfants, fonctionne en complément d'une présence scolaire aménagée et dans l'attente d'une intégration en établissement spécialisé. Au total, 128 enfants ont pu y être accueillis en un peu plus de deux ans. En outre, les mercredis et lors des périodes de vacances, il devient un centre de loisirs inclusif. Ce dispositif, géré par des professionnels et des bénévoles, donne entière satisfaction aux enfants ainsi qu'à leurs familles. Malheureusement, sa continuité est menacée au-delà du 31 décembre prochain, car une partie car une partie des financements exceptionnels qui ont permis sa création ne seraient pas renouvelés. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, quels financements pourraient être accordés pour pérenniser ce type d'initiative qui fait évoluer favorablement la prise en charge du handicap,

Pour autant, avec un démarrage en janvier 2020, le travail sur le répit a été percuté par la crise sanitaire- vous l'avez rappelé. En réaction, les porteurs de projets et les financeurs ont développé des réponses aux situations créées par l'interruption des accueils de jour ou des prises en charge en libéral. la crise sanitaire a été l'occasion pour tous les acteurs de faire preuve de créativité et d'agilité dans l'organisation, l'autorisation et le financement de solutions de répit. Il faut saluer ce travail et ces résultats. Certaines solutions avaient vocation à répondre spécifiquement aux situations créées par le confinement. D'autres peuvent répondre à des besoins pérennes. Le dispositif « On Prend Le Relais ! » a été créé dans ce contexte, et continue de répondre aux besoins d'accueil de loisirs des enfants en situation de handicap sur votre territoire. À ce titre, il bénéficie d'un financement par la caisse d'allocations familiales (CAF). J'ai demandé à mes services de regarder attentivement la situation de ce dispositif auprès de

qui sera lancée à compter de 2023. L'effort sur le répit sera poursuivi en réinterrogeant le format des solutions proposées aux personnes, leur cadre juridique et leur financement. Cette amélioration s'appuiera entre autres sur des travaux nationaux, la Haute Autorité de santé (HAS). Il nous appartiendra de rester attentifs à l'ensemble des expériences menées sur le terrain qui apportent des réponses concrètes aux parents. L'accueil périscolaire et de loisirs pour les enfants en situation de handicap sera une priorité et devra être renforcé.

pour l'ensemble de la région. Pourtant, les élus de l'Yonne, les personnels de santé et les habitants souhaitent maintenir cette présence en mutualisant les centres d'appels du 15 et du 18. Exact ! Cependant, le projet n'avance pas, l'ARS ne communique pas et le flou perdure. Ainsi, madame la ministre, ma question est particulièrement simple : le Gouvernement et l'ARS sont-ils enfin prêts à s'engager dans une démarche de concertation et de travail avec tous les acteurs locaux afin de faire aboutir ce projet ?

de Bourgogne-Franche-Comté a mis en lumière une très forte hétérogénéité dans l'organisation des centres de réception et de régulation des appels (CRRA) d'aide médicale urgente. Une problématique d'effectifs a également été identifiée, entraînant dans certains départements des déficits caractérisés.

Dans le cadre de cet audit, l'ensemble des acteurs concernés- professionnels, élus locaux, parties prenantes -, y compris ceux du département de l'Yonne, ont eu l'occasion de faire entendre leur voix. Plus de soixante-dix personnes ont été auditionnées. Cette évaluation a montré qu'un certain nombre d'objectifs assignés au regroupement ont bien été atteints. Elle a également permis d'identifier des pistes pour renforcer encore la solidarité et la coopération entre les acteurs. L'ARS a rappelé que cette évaluation constituait un préalable à toute nouvelle évolution de l'organisation des autres centres 15 de la région. Ainsi, en août 2022, il a été proposé aux acteurs de l'Yonne de confronter les résultats de l'évaluation à l'examen spécifique de leur département. Cette démarche alimentera les travaux de révision du projet régional de santé, qui doivent aboutir à l'automne 2023. Elle devra intégrer une une logique de sécurisation et d'entraide entre les CRRA et le 15. Cette révision s'effectuera dans le cadre d'une large concertation avec les acteurs des territoires, à laquelle vous serez associée et dont il vous sera rendu compte.

La reconstruction de ce CHU a été annoncée en 2018. Ce projet ambitieux, porté par l'État, offrira un outil et un cadre de soins modernes aux soignants et aux patients. de 2022, la première phase de cette reconstruction s'achèvera ; pour la seconde phase, ce sera en 2026. Néanmoins, le devenir de l'actuelle « Tour de Nacre » du CHU, inaugurée en 1975 par Simone Veil, reste à régler. En effet, le bâtiment a été conçu à une période où l'isolation et le cloisonnement faisaient la part belle à l'amiante pour les constructions. Un rapport de la chambre régionale des comptes soulignait en 2019 que le bâtiment présentait « un niveau particulièrement élevé d'amiante Il relevait ainsi que « la structure actuelle ne garantit pas la sauvegarde du bâtiment et des personnes en cas d'incendie généralisé ». Sa structure empêchant de surcroît « tous travaux de rénovation à des coûts acceptables »,

et le seul désamiantage. À quelques semaines de la fin de la première phase de la reconstruction du CHU de Caen et de l'inauguration des premiers pavillons, la question de l'avenir de cette tour devient plus que pressante.

Pas moins de 400 millions d'euros de crédits de soutien de l'État sont consacrés à ce projet, soit plus de 70 % du plan de financement. Ce projet s'inscrit en deux phases. Certains bâtiments-

En parallèle, sur le bâtiment actuel de la Tour de Nacre, d'importants travaux de mise en sécurité ont été entrepris par le CHU de Caen, avec le soutien financier de l'ARS de Normandie, portant notamment sur la sécurité incendie et le risque amiante. Ces travaux ont permis au CHU de considérablement améliorer sa capacité de réponse au risque incendie. Par ailleurs, les secteurs qui présentaient un risque d'exploitation lié à la présence d'amiante ont été traités et sécurisés. Tous les matériaux contenant de l'amiante et à risque, en cas d'usure, ont été retirés. Les équipes techniques du CHU sont exemplaires dans la surveillance environnementale du bâtiment et la gestion de l'ensemble des aspects liés à ce sujet. À la livraison du nouveau CHU, la Tour de Nacre n'accueillera plus de public. Un plan de continuité sera mis en oeuvre pour assurer la maintenance incompressible et la sûreté des installations.

Mais les fractures territoriales demeurent et s'exacerbent. L'an dernier, un chiffre avait marqué les esprits : on vit en moyenne deux années de moins à la campagne qu'en ville. Loin de lutter contre ces inégalités indignes de notre République, le Gouvernement les alimente. Dans une mission flash de juin dernier sur les urgences et soins non programmés, il était indiqué qu'« une équipe d'intervention hospitalière ne pouvait être composée que d'une équipe paramédicale dans une logique d'adaptation pragmatique ». C'est le cas dans l'Oise, où les habitants du Noyonnais se verront bientôt envoyer des ambulances sans médecin. Doit-on en conclure que « l'adaptation pragmatique » à la pénurie de soignants, c'est tout simplement se passer d'eux ? C'est le sens de la réforme engagée par la direction du centre hospitalier intercommunal

de la voix de nombreux élus locaux, vent debout face à une mesure qui pénalisera avant tout les communes rurales déjà éprouvées, sinon accablées, par le manque de praticiens. Je vous remettrai d'ailleurs une motion du conseil départemental de l'Oise et une pétition d'une soixantaine de maires qui vous feront prendre la mesure de cette opposition résolue et quasi unanime. Le Gouvernement envoie un signal plus qu'inquiétant à l'égard de nos territoires les plus fragilisés. Ils paieront le prix de la technocratisation des politiques de santé, où les agences régionales de santé décideront seules de la généralisation de ces équipes d'urgence paramédicalisées. paramédicalisées. En juin 2021, le syndicat des médecins libéraux alertait déjà sur les risques que font peser ces protocoles hybrides sur la responsabilité professionnelle des soignants et la sécurité des patients. Alors, madame la ministre, comptez-vous renoncer à cette réforme du Smur, qui met en péril le principe le plus fondamental de notre sécurité sociale, celui de l'égal accès aux soins ?

dite « équipe paramédicale de médecine d'urgence », a été expérimentée cet été, en particulier dans le département de la Sarthe. Les équipes ont donné totale satisfaction, intervenant soit seules, soit en avant-coureurs du Smur, en lien étroit avec le médecin régulateur du

Face aux difficultés rencontrées pour faire fonctionner ces trois lignes, faute de ressources médicales suffisantes, la direction a pris la décision de mettre en place cette organisation en équipe paramédicale à Noyon. Cette organisation permet de maintenir une ressource médicale aux urgences de Noyon, et donc d'assurer la prise en charge des patients sur ce site. Elle garantit la présence d'un professionnel paramédical formé, en jonction, le cas échéant, avec un vecteur médicalisé. Elle permet également de consolider les urgences de Compiègne. Les formations des infirmiers par le Samu de l'Oise sont en cours, avec des sorties « doublées et supervisées » par un médecin. Le fonctionnement de ce dispositif fera l'objet d'une évaluation et d'une attention toute particulière de l'ARS des Hauts-de-France, et il en sera bien entendu rendu compte aux élus du territoire.

Cette dernière rayonne sur un bassin de vie pour le moins étendu, jusqu'aux portes d'Alès, et surtout à travers les montagnes cévenoles. Je le précise car, par voie de conséquence,

La fermeture de cette maternité, qui sera donc effective dès le 20 décembre prochain, imposera aux patientes un trajet de plus d'une heure, voire de deux heures, pour rejoindre Nîmes ou Montpellier. Elle fait donc courir un risque aux enfants et à leurs mères.

Le plus rageant, madame la ministre, c'est la raison de cette fermeture ! Ce service restera fermé, non par manque de fréquentation, mais le temps de recruter des gynécologues, des anesthésistes et des pédiatres ; nous en sommes donc là dans la France de 2022 J'ai d'ailleurs appris dans la presse que le groupe Cap Santé avait publié des offres d'emploi partout en France, et même à l'étranger, avec des niveaux de rémunération comparables à ceux qui se pratiquent partout.

mais d'une suspension de l'activité pour une durée indéterminée, le temps de reconstituer une équipe soignante suffisante. L'autorisation de gynécologie-obstétrique est maintenue à la clinique et sera inscrite au plan régional de santé Afin d'assurer le maintien des autres activités- suivi pré-et post-natal, préparation à l'accouchement, suivi des bébés et des enfants -, un centre périnatal de proximité pourra être mis en place, en associant les professionnels de la clinique et les professionnels libéraux, sous la coordination des (CHU) de Montpellier et de Nîmes. L'activité d'IVG sera maintenue. Il faut également souligner que les difficultés spécifiques de la maternité sont à dissocier des efforts faits dans les autres services de la clinique. d'urgence et de réanimation (Smur), la chirurgie et la médecine doivent être renforcés et développés dans le cadre de la reconstruction de la clinique, dont le projet a été acté et soutenu par l'ARS d'Occitanie. On peut, à ce titre, mentionner l'autorisation d'un nouvel appareil IRM à la clinique, qui est une preuve tangible de l'investissement des acteurs et de l'État dans l'avenir du site de Ganges. Nous devons

à l'hôtel, la fin des « sorties sèches » de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à l'âge de 18 ans, ainsi qu'une meilleure protection contre les violences. Si ces progrès sont à saluer, les acteurs de ce secteur, auxquels je rends hommage pour leur investissement et leur dévouement, considèrent qu'il faut aller plus loin. Alors que les départements constituent la pierre angulaire de la protection de l'enfance, il existe une grande disparité des pratiques en fonction des territoires, qui résulte d'un manque de pilotage à l'échelle nationale. Selon le département dans lequel ils se trouvent, les enfants protégés ne sont pas pris en charge de la même manière. Il est donc important que les départements bénéficient d'un plus grand soutien de l'État, notamment sur le plan financier, pour exercer pleinement leurs missions sociales. Notre politique de protection de l'enfance est insuffisante en matière de repérage et de prise en charge des troubles psychiatriques. Compte tenu de leur parcours de vie, de nombreux enfants protégés sont pourtant en souffrance. Dans son rapport annuel consacré aux droits de l'enfant, la Défenseure des droits a alerté sur l'urgence de mieux protéger la santé mentale des enfants les plus fragiles, précisant que les besoins en soins de pédopsychiatrie avaient plus que doublé en vingt ans. Alors que certains enfants doivent parfois attendre plus d'un an pour être pris en charge, les professionnels de l'aide à l'enfance réclament un véritable « plan Marshall pour la pédopsychiatrie. Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour garantir pleinement l'intérêt supérieur des enfants protégés ?

le Président de la République a souhaité faire de l'enfance et de sa protection un des sujets prioritaires pour les prochaines années. Dans votre question, vous avez cité la loi du 7 février 2022 : si bien des choses ont été faites au cours du précédent quinquennat, il reste encore beaucoup à faire. La secrétaire d'État Charlotte Caubel est pleinement mobilisée pour mettre en oeuvre la loi de 2022. Plusieurs décrets ont déjà été publiés : je pense notamment à celui relatif aux jeunes majeurs et à celui sur la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux. D'ici à la fin de l'année, d'autres le seront, comme celui sur l'interdiction totale en 2024 de l'hébergement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs. Nous travaillons également à mieux accompagner les départements, une orientation à laquelle- je Nous réfléchissons actuellement avec eux à la future vague de contractualisation, à laquelle nous souhaiterions associer les ministères de l'éducation et de la justice. Nous travaillons aussi au renforcement de la coordination des acteurs de terrain- est forte en la matière -grâce à la mise en place des conseils départementaux de la protection de l'enfance. Enfin, la Première ministre a réuni la semaine dernière le premier comité interministériel à l'enfance. Avec les ministres concernés, nous avons déterminé une quarantaine de mesures structurées autour des axes prioritaires : lutter contre les violences faites aux enfants, garantir l'égalité des chances

Face aux arrêts maladie, aux difficultés de recrutement et à l'épuisement des personnels, des mesures ont été prises pour renvoyer vers d'autres structures les cas les plus graves. Mais il faut souligner que ces mesures se sont heurtées à plusieurs écueils majeurs. En effet, la médecine de ville, elle aussi exsangue, ne peut prendre le relais aux solutions numériques de renvoi vers des systèmes de cartographie des soins, elles sont inadaptées aux personnes en situation d'illectronisme. Ces situations ne sont que provisoires, et vous comprendrez que les élus souhaiteraient avoir une véritable stratégie d'accueil durable des patients en situation d'urgence dans le département, de jour comme de nuit. Au-delà de la situation de Manosque, qui demeure très fragile, notamment pendant les périodes d'afflux touristique, c'est toute l'organisation de l'offre hospitalière du département qui ne cesse d'évoluer. Les périodes très longues de fermeture des urgences de son hôpital ont d'ailleurs affecté les habitudes prises par les patients de celui-ci.

Madame la ministre, la proximité constitue un enjeu majeur d'efficacité de la médecine d'urgence, avec la connaissance fine de l'environnement et des acteurs concernés.

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, les difficultés rencontrées par les urgences du site de Manosque s'inscrivent aussi dans un contexte national de manque d'urgentistes, qui exacerbe La situation des urgences fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement, comme en témoignent les mesures prises cet été et mises en place grâce à la mission du ministre de la santé François Braun.

le renforcement de la médecine de ville, qui va de pair avec le réflexe du recours au 15 pour éviter des passages injustifiés aux urgences. Au niveau local, les tensions sur le service d'accueil des urgences de Manosque

Pour combler le manque de personnels, des appels à candidatures ont été lancés et la prime de solidarité territoriale a été majorée. La fusion, un temps évoquée, du Samu des Alpes-de-Haute-Provence avec celui de Hautes-Alpes n'est plus à l'ordre du jour. L'enjeu est d'encourager les synergies et les mutualisations, par exemple en faisant opérer la régulation certaines nuits depuis le centre 15 de Digne et les autres depuis Gap. Par ailleurs, l'ARS soutient le déploiement de dispositifs innovants d'aide médicale d'urgence dans les territoires difficiles d'accès pour le Smur.